Je vous rappelle que, pour cette mission, la conférence des présidents a fixé la durée maximum de la discussion à deux heures trente. En conséquence, si nous n'avions pas terminé l'examen de cette mission à quinze celui-ci se poursuivrait à la fin des missions de cette semaine ou la semaine prochaine, et nous passerions à l'examen de la mission « Sport, jeunesse et vie associative ». La parole est à M. le président de la commission des finances.

d'autorisations d'engagement constituent la première tranche de cette ambition. À ces quatorze avions s'ajoutent deux avions supplémentaires en cours d'acquisition dans le cadre du mécanisme de protection civile de l'Union européenne Au total, en intégrant les appareils financés par le programme européen, la flotte aérienne de la sécurité civile sera ainsi composée de seize avions amphibies bombardiers d'eau.

devaient être opérationnels à l'horizon 2027. Cependant, il semble que la chaîne de fabrication vienne juste d'être lancée et, d'après les avis de personnes spécialisées, il sera quasiment impossible de respecter les délais avancés, ne serait-ce que la livraison de deux appareils avant 2027.

particulièrement importantes de l'été 2022 et dans la perspective d'événements hors normes, il est apparu que nous devions disposer de moyens humains suffisants. Il paraît indispensable de favoriser l'engagement de l'ensemble des sapeurs-pompiers. Cet amendement vise donc, d'une part, à financer vise donc, d'une part, à financer les remboursements aux services d'incendie et de secours liés à la création d'une indemnité de mobilisation opérationnelle exceptionnelle au profit des sapeurs-pompiers professionnels

Enfin, fort du retour d'expérience de la saison de feux de l'année 2022, le Gouvernement entend renforcer les vecteurs aériens de l'année 2023 par l'augmentation du nombre d'hélicoptères bombardiers d'eau en location, ce

de la gendarmerie et de la police nationales et sur la création de 200 brigades supplémentaires sur un effectif existant de 3 200 brigades.

on s'aperçoit que les seules mesures catégorielles concernant le titre 2, c'est-à-dire les mesures de personnel de gendarmerie, sont d'un montant supérieur à l'investissement nécessaire dans l'immobilier.

Cet amendement vise à augmenter les crédits affectés aux moyens nationaux de la sécurité civile, afin de permettre l'achat et l'entretien de nouveaux hélicoptères en vue d'assurer une meilleure couverture du territoire métropolitain, en transférant 30 millions d'euros de l'action n° 04 du programme 152 vers l'action n° 12 du programme 161. Le renouvellement de l'extension de la flotte d'hélicoptères de la sécurité civile a déjà été acté dans le cadre de la Lopmi et se traduira par la livraison de trente-six appareils. Ainsi, la flotte devrait être portée à quarante hélicoptères, ce qui correspond à l'objectif fixé par le ministère de l'intérieur.

La question de la couverture territoriale de la flotte d'hélicoptères de secours ne concerne donc pas uniquement les appareils de la sécurité civile et doit faire l'objet d'une réflexion à l'échelon interministériel. La commission émet un avis défavorable sur cet

En revanche, il est prévu un pacte capacitaire qui viserait à renforcer les moyens de différents Sdis. Ce premier pas du Gouvernement est intéressant,

qui constituent des outils majeurs de modernisation de la réponse opérationnelle de la sécurité civile, ainsi que la garantie d'une couverture territoriale

a surtout développé les brigades vertes ou la gendarmerie verte. Nous suivons l'évolution de cette initiative. En revanche, il me semble peu opportun de créer un programme budgétaire uniquement sur ce sujet.

la Défenseure des droits, en charge de la déontologie des forces de l'ordre.

C'est un amendement ciblé ... Dans de nombreux endroits, l'accueil des victimes, d'une manière générale, n'est pas toujours très satisfaisant.

Présents dans certaines grandes villes de France, ils sont chargés de recevoir les plaintes et de traiter les procédures liées à l'homophobie et à la transphobie. Quel est l'avis de la commission

justifié que des crédits de l'État soient consacrés à l'acquisition d'engins de lutte anti-incendie au bénéfice d'un seul département.

par les autorités de sécurité publique ouvre la voie à l'expérimentation pour les sapeurs-pompiers professionnels, volontaires et militaires, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et les marins-pompiers de Marseille. La loi du 25 novembre 2021

obligatoires aux tirs et aux pratiques professionnelles en intervention prévus chaque année pour garantir le niveau d'aptitude des agents ne sont pas systématiquement respectés dans la pratique. Cet amendement vise à combler cette lacune.

émet un avis défavorable, bien que je partage le constat sur la nécessité de renforcer la prévention, notamment en matière de lutte contre les feux. Cet amendement ne semble pas apporter une solution satisfaisante à cette question, qui ne saurait être réglée par un abondement de crédits budgétaires. La prévention des feux de forêt doit s'inscrire dans le cadre d'une stratégie multidimensionnelle dépassant les seuls enjeux financiers. Je pense notamment aux obligations légales de débroussaillement ou à la définition d'une ou à la définition d'une stratégie efficace de prépositionnement des moyens aériens de lutte contre les feux de forêt. Quel est l'avis que soutenir l'effort de développement de l'offre de services de Météo-France et de l'ONF pour une meilleure connaissance et une meilleure prévention des risques de feux de forêt. Néanmoins, la prévention du risque et sa connaissance sont de la

L'indicateur modifié permettra de mieux évaluer le poids des activités de patrouille de voie publique dans l'activité totale de la police et de la gendarmerie nationales.

sous la labellisation « nombre d'heures de patrouille de voie publique ». L'indicateur modifié permettra de mieux évaluer le poids des activités de patrouille de voie publique dans l'activité totale de la police et de la gendarmerie nationales. Il est plus significatif avec cette mise en perspective, dans la mesure où le simple décompte des heures de patrouille ne permet pas de déterminer quel est le poids de cette activité pour les forces de sécurité intérieure.

l'avis du Gouvernement.

mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés entendait permettre le cumul des revenus des pensions de retraite avec ceux d'une activité exercée dans le secteur privé.

M. Patrick Kanner, président du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, demande, dans le cadre de l'ordre du jour réservé à son groupe du mercredi 7 décembre, que la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à lutter contre la précarité des accompagnants d'élèves en situation de handicap et des assistants d'éducation soit examinée en remplacement de la proposition de loi relative à la titularisation des accompagnants d'élèves en situation de handicap et des assistants d'éducation, présentée par Mme Sylvie Robert et plusieurs de ses collègues. Ces deux propositions de loi contenant des dispositions quasiment identiques, nous pourrions, en accord avec la commission de la culture, déroger à titre tout à fait exceptionnel au délai de six semaines prévu entre la demande d'inscription à l'ordre du jour et l'examen en séance publique. Y a-t-il des observations ? ... Il en est ainsi décidé.

d'État, mes chers collègues, cette année, la mission « Sport, jeunesse et vie associative » ne comporte aucune mesure nouvelle de grande ampleur, mais elle voit ses dispositifs existants renforcés. La mission bénéficie ainsi d'une hausse notable de ses crédits, de 5,8 %, soit exactement 100 millions d'euros de plus que l'année dernière. Avant l'examen de la mission,

Selon un sondage de l'institut Odoxa datant de la rentrée, un quart des Français auraient renoncé à pratiquer un sport à cause de l'inflation. Quant aux associations, en raison de leur public cible, elles ont souvent des réticences à augmenter leur tarif, ce qui peut aggraver leurs difficultés financières. La situation impose donc de s'interroger sur l'efficacité des dispositifs d'aides aux associations et à la pratique sportive. Le Pass'Sport, dispositif ciblé sur les ménages modestes, a été reconduit en 2023, pour un budget de 100 millions d'euros, identique à celui de l'année dernière. Si c'est un outil intéressant, il souffre d'un non-recours important : seuls 18,3 % des jeunes éligibles ont formulé une demande. L'Agence nationale du sport (ANS) bénéficie d'un rehaussement de 7,5 % de sa subvention, qui atteint 264,7 millions d'euros. Le renforcement de ses moyens doit être l'occasion de mener une réflexion sur la gouvernance : la « nouvelle gouvernance du sport » doit laisser une place importante aux acteurs du sport, mais elle ne doit surtout surtout pas être synonyme d'un désengagement de l'État. Une gouvernance solide est essentielle alors que les jeux Olympiques et Paralympiques se profilent. Les tensions sur le marché de l'énergie et sur le marché des matières premières ont déjà des conséquences importantes sur la préparation de ces événements. Selon la direction des sports, le besoin de financement supplémentaire pour la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo) est évalué à 143 millions d'euros, dont les deux tiers seront pris en charge par l'État. Au-delà du seul budget de la Solideo, j'évoquerai les enjeux financiers plus larges de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques.

Je conclurai mon propos en évoquant le soutien aux associations et les politiques d'engagement de la jeunesse. Le compte d'engagement citoyen (CEC), qui voit ses crédits diminuer pour 2023, ne tient pas encore ses promesses. Alors que le nombre d'ayants droit était estimé à 400 000 à la fin de l'année 2021, seuls 3 192 dossiers ont été validés. Je pense qu'il s'agit d'une idée intéressante pour valoriser l'engagement bénévole, mais le fonctionnement du dispositif doit être revu. Le service national universel (SNU) continue sa montée en charge. Son budget est désormais de 140 millions d'euros, l'objectif pour 2023 étant que 64 000 jeunes accomplissent ce service, contre 50 000 cette année.

Les centres pouvant accueillir les jeunes effectuant le séjour de cohésion sont en nombre limité, il est difficile de recruter des encadrants et la construction d'une administration du service national universel prend du temps. J'ai pu constater l'engagement des équipes pour offrir aux jeunes un séjour de qualité, mais je reste sceptique à la fois sur l'opportunité et la faisabilité de la généralisation du service national universel. Au nom de la commission des finances, je mène un contrôle budgétaire sur le SNU et nous rendrons nos conclusions durant le premier semestre de 2023. Le service civique bénéficie, lui, de 518,8 millions d'euros en 2023, ce qui représente une augmentation de 20 millions d'euros par rapport à 2022, mais une diminution de crédits par rapport au plan de relance. J'ai souvent exprimé mes réserves sur le recours au service civique dans le cadre du plan de relance. Plutôt qu'une politique de stop-and-go, je défends encore et toujours une montée en charge progressive du dispositif, qui permettrait de mettre en place des missions plus intéressantes et valorisantes, et de rassurer les opérateurs. Le budget du service civique présenté dans le projet de loi de finances m'apparaît à cet égard satisfaisant. Au regard de ces éléments, la commission des finances a décidé de proposer au Sénat d'adopter sans modification les crédits de la mission « Sport, jeunesse et vie associative ». La parole est à M. le rapporteur

madame la ministre, mesdames les secrétaires d'État, mes chers collègues, l'examen des crédits consacrés au sport conduit à des conclusions différentes, selon que l'on regarde l'année 2023 ou les années 2024 et 2025. À court terme, on peut estimer que le monde du sport a plutôt bien résisté à la crise sanitaire. Le projet de loi de finances pour 2023 reconduit plusieurs dispositifs utiles, comme le Pass'Sport ou le plan en faveur du développement des équipements de proximité.

Hormis la question des taxes affectées, sur laquelle nous reviendrons au cours de notre débat, on peut saluer la hausse de 3 % des crédits consacrés au sport, même si cette augmentation signifie en réalité une baisse en euros constants, compte tenu de l'inflation attendue en 2023. À moyen terme, en revanche, les nuages semblent s'amonceler sur l'horizon du sport. Les crédits du plan de relance mobilisés pour améliorer l'isolation thermique de certains équipements sportifs n'ont pas été reconduits, alors que sévit une crise énergétique sans précédent. La discussion du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 a révélé que le Gouvernement prévoyait de baisser les crédits consacrés au sport à l'issue des jeux Olympiques et Paralympiques.

S'agissant des infrastructures olympiques, la Solideo tient son calendrier et son budget en euros constants, même si elle a besoin de 150 millions d'euros pour faire face à l'inflation, dont un tiers serait à la charge des collectivités territoriales.

Nous constatons que les hypothèses sur lesquelles les jeux Olympiques et Paralympiques ont été pensés ne tiennent plus aujourd'hui, et ce pour des raisons indépendantes de la volonté des organisateurs. Mais, au-delà de ce rendez-vous olympique, la question de l'avenir de notre ambition pour le sport est posée. Nous aurons bien un rendez-vous en 2024, madame la ministre, comme vous l'avez indiqué en commission. À cette fin, nous avons besoin d'y voir clair sur le financement du sport dans les années à venir, ce qui passe, selon moi, par trois priorités : la réouverture du débat sur l'attribution au sport de la totalité du produit des trois taxes affectées ou la recherche d'un financement alternatif aux crédits extrabudgétaires actuels le lancement d'un grand plan de rénovation de nos équipements structurants et locaux, notamment pour répondre à la crise de l'énergie ; l'accélération de la mise en oeuvre de la gouvernance territoriale de l'ANS, qui n'est pas encore pleinement opérationnelle.

madame la ministre, mesdames les secrétaires d'État, mes chers collègues, la commission de la culture a examiné le programme 163, « Jeunesse et vie associative », doté pour 2023 de 837 millions d'euros, soit une augmentation de 65 millions d'euros par rapport à 2022. Toutefois, cette augmentation s'explique en grande partie par la montée en charge du service national universel, dont les crédits dédiés augmentent encore de 30 millions d'euros, malgré les nombreuses réserves émises depuis sa création.

Pour l'encadrement des jeunes, le recours massif au contrat d'engagement éducatif (CEE) n'est en aucun cas adapté aux particularités du dispositif. Par ailleurs, encore trop peu de jeunes réalisent les missions d'intérêt général de la phase 2.

ils sont en augmentation de 20 millions d'euros. Cette hausse, bienvenue, doit être nuancée par l'arrêt du financement des missions lancées dans le cadre du plan de relance, qui représentaient environ 200 millions d'euros. Pourtant, le service civique a fait ses preuves et démontre, chaque année davantage, son efficacité en termes d'accompagnement et d'insertion des jeunes. Dans le même temps, l'effort en faveur de la jeunesse et de l'éducation populaire, visible notamment au travers des mesures issues des Assises de l'animation, doit être souligné.

candidats. La rentrée scolaire de 2021 a effectivement été marquée par de grandes difficultés dans le secteur des accueils collectifs de mineurs, parmi lesquels les colonies de vacances. Face à l'ampleur des besoins, il faut redonner aux jeunes l'envie de s'investir davantage dans ces secteurs en crise. Enfin, j'évoquerai la diminution des crédits en faveur du développement de la vie associative. Plus que jamais, il m'apparaît essentiel de renforcer le soutien aux associations, qui peinent à retrouver leur dynamisme d'avant-crise. L'activité bénévole demeure trop peu valorisée, et les dispositifs à destination des bénévoles mal connus et peu lisibles. Cette fragilisation du tissu associatif, accentuée par l'impact de la crise énergétique sur les activités associatives, est particulièrement préoccupante pour la survie des petites associations.

Comme vous pouvez le constater, mes chers collègues, la répartition des crédits supplémentaires en faveur de la jeunesse et de la vie associative pose question. C'est pourquoi la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a décidé de s'abstenir sur l'adoption des crédits du programme 163. Mes chers

pour atteindre 1 822,2 millions d'euros en crédits de paiement. Cette hausse se concentre principalement sur les politiques dédiées à l'engagement des jeunes, la poursuite du plan en faveur des équipements sportifs de proximité et, enfin, l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Les crédits consacrés au sport devraient augmenter de près de 3 %, pour atteindre 818,3 millions d'euros. Je salue la poursuite du plan consacré aux équipements de proximité, 100 millions d'euros de nouveaux crédits étant prévus en 2023 et 2024, ainsi que la reconduction du Pass'Sport pour 100 millions d'euros en 2023. Ce Pass bénéficiera à de nouveaux publics, puisque les étudiants boursiers et les jeunes bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) y ont désormais accès. C'est une bonne chose, tant le sport véhicule des valeurs essentielles, mais les crédits restent trop peu consommés. Le taux de recours au Pass est seulement de 18 %. Il est essentiel de continuer à faire la promotion de ce dispositif sur l'ensemble du territoire, pour qu'il bénéficie au plus grand nombre. Je regrette l'insuffisante prise en compte de la dégradation de la situation économique. La crise énergétique a dès à présent des conséquences sur les familles, les collectivités territoriales et l'ensemble des acteurs du secteur. Les crédits du plan de relance concernant l'accompagnement à la rénovation thermique des bâtiments dédiés à la pratique sportive n'ont pas été reconduits, tandis que les élus locaux font face à l'explosion des coûts de fonctionnement. Concernant les jeux Olympiques et Paralympiques, les crédits accordés sont globalement stables, atteignant 294,9 millions d'euros. L'éventualité de pénuries de matériaux de construction représente un risque supplémentaire. Nous serons attentifs à la question du dépassement budgétaire, tout comme au respect du calendrier par la Solideo. Le sport est parfois le meilleur des remèdes. Notre groupe est favorable à la poursuite d'une réflexion sur la prise en charge par la solidarité nationale de séances d'activité sportive dans le cadre de nos politiques de prévention de la perte d'autonomie.

les crédits destinés à la vie associative sont en baisse- je le regrette. L'écosystème associatif, composé principalement de petites structures, reste particulièrement fragilisé par la crise sanitaire. Après la période de repli sur soi que nous avons connue pendant la crise de la covid-19, il faut redonner du souffle au monde associatif, qui souffre cruellement. Pour la jeunesse, le projet de loi de finances fait état d'une progression de 20 millions d'euros des crédits dédiés au service civique, soit une hausse de 15 %. Je salue la poursuite de cette dynamique, particulièrement visible en milieu rural. En revanche, la baisse drastique du nombre de candidats au Bafa, malgré les aides mises en place, doit nous alerter. De son côté, le service national universel devait initialement concerner 400 000 jeunes au cours de l'année 2022. En réalité, il n'y avait que 50 000 places disponibles, qui n'ont pas toutes été pourvues, malgré la qualité des encadrements. Ce dispositif est une bonne idée, mais il peine à se hisser à la hauteur de ses ambitions. En 2023, le PLF lui accorde 140 millions d'euros, soit une hausse de 30 %. Avant d'annoncer sa généralisation, il faut s'assurer que la prise en charge sera réelle, dans l'ensemble des territoires, et qu'il ne s'agit pas simplement d'effets d'annonce. Pour ce qui est des jeux Olympiques et Paralympiques, il est essentiel de favoriser des retombées concrètes sur tout le territoire national et de généraliser la pratique sportive, pour les jeunes, pour la santé et l'inclusion sociale des Français. Pour gagner, nous devons rehausser notre niveau de jeu, à nouveau partout sur le territoire, et profiter de cet événement d'ampleur pour faire de la France une nation sportive avant, pendant et après cette échéance.

mais, ne nous y trompons pas, cette architecture budgétaire large ne doit rien au hasard. Elle traduit une volonté politique claire et assumée d'empêcher l'émergence d'une réelle politique d'éducation populaire tournée vers l'émancipation. Disons-le clairement,

Pour nous, c'est un dispositif inutile, fondé sur une nostalgie surannée du service militaire, un dispositif au fumet autoritaire, pensé pour faire « rentrer la jeunesse dans le rang », la faire obéir, la faire saluer au garde-à-vous, y compris des responsables civils. Un dangereux mélange des genres La liste des scandales entourant le SNU ne cesse de s'allonger au fil des mois : malaises de jeunes laissés en plein soleil, brimades et punitions physiques collectives, désorganisation des convocations et, même, atelier de menottage en lien avec la police nationale.

ensuite de cette discussion budgétaire pour relayer les craintes du mouvement associatif. Certaines, qui concernaient une mise au pas des associations les plus militantes, s'étaient exprimées au moment de l'examen de la loi, dite Séparatisme,

Les annonces concernant la mobilisation du fonds vert pour rénover les équipements devraient nous rassurer. Mais, comme tous les ministres semblent vouloir se servir dans ce fonds, nous sommes très dubitatifs sur les montants qui seront réellement J'ai été surpris- mais pas vraiment étonné, tant c'est le cas dans toutes les missions budgétaires -de l'absence du mot climat dans la présentation du programme « Sport ». J'ai compris pourquoi lorsque nous avons eu confirmation de la présence de notre ministre des sports à la Coupe du monde de football organisée au Qatar, et donc de la caution apportée, par sa présence, à l'aberration, pour ne pas dire à la bombe la bombe climatique, que constitue cet événement. C'est toujours le même déni gouvernemental sur les questions climatiques, que nous connaissons depuis cinq ans ! Pourtant, le changement climatique aura des conséquences dramatiques sur les pratiques sportives, les stations de ski, les installations littorales, le sport en extérieur et en plein été. De tout cela, il n'est pas prévu de débattre aujourd'hui, à la lecture de ce budget, et c'est pourquoi nous aborderons ce sujet par voie d'amendement. J'évoquerai un dernier point, et pas des moindres tant il constitue presque l'horizon unique de la politique sportive française des prochaines armées : les jeux et Paralympiques de 2024. Le budget poursuit une trajectoire financière qui, sans surprise, commence à déraper- mais tout cela était prévu de longue date. Je dois en revanche me faire ici l'écho des inquiétudes relatives à l'annulation possible des festivals en 2024, qui plonge dans l'insécurité de nombreuses entreprises culturelles, peinant déjà à relever la tête après la pandémie de covid-19. Le risque d'opposer sport et culture est grand. La fête des jeux Olympiques et Paralympiques ne doit pas être gâchée par une saison de festivals annulée de plus. Il est donc nécessaire de mieux dimensionner la mobilisation de nos forces de sécurité pour que saison culturelle et jeux puissent se dérouler en harmonie. Pour conclure, s'agissant du sport, nous constatons la faiblesse des ambitions climatiques ; s'agissant de la jeunesse, nous refusons la mise au pas annoncée

En témoigne l'augmentation de 5,1 % des crédits de la mission « Sport, jeunesse et vie associative », qui atteignent 1,82 milliard d'euros en crédits de paiement. Ces moyens financiers permettent de poursuivre l'accès des jeunes à la pratique sportive, avec le Pass'Sport, un dispositif pertinent qui porte ses fruits et que nous devons amplifier. Je me réjouis donc de son extension à de nouveaux publics : les étudiants jusqu'à 28 ans révolus bénéficiant d'une bourse sur critères sociaux de l'enseignement supérieur et les jeunes bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés. Je salue également le déploiement des parcours sport-santé de proximité sur les territoires, sans oublier les 100 millions d'euros destinés au financement du programme des 5 000 équipements sportifs de proximité, soit 200 millions d'euros sur deux ans pour développer la pratique sportive sur tout le territoire national, l'objectif étant d'atteindre trois millions de nouveaux

proximité. Pour garder cette proximité- je profite de l'occasion pour vous interroger, madame la ministre -, le zonage ne pourrait-il pas être retravaillé afin d'éviter l'exclusion de certains territoires, qui ne sont situés ni dans les zones de revitalisation rurale ni dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ? positif pour l'engagement de la jeunesse. Dans une société divisée, où de nombreux jeunes sont en quête de repères, je pense que le service national universel mérite Je suis donc plus qu'étonné de voir le nombre d'amendements déposés pour réduire les moyens financiers qui lui sont dédiés. Les auteurs de ces amendements considèrent-ils que le service national universel ne mérite pas de bénéficier de bénéficier d'une enveloppe supplémentaire de 30 millions d'euros ? Je pense au contraire, mes chers collègues, que nous ne dépenserons jamais assez d'argent pour l'engagement de notre jeunesse au service de l'intérêt général et des valeurs de la République. Enfin, je ne peux terminer sans revenir un instant sur sur les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Les crédits du programme dédié diminuent de 0,7 %, ce qui démontre que la trajectoire budgétaire a été anticipée et demeure maîtrisée. Certes, le comité d'organisation vient d'annoncer cette semaine un coût supplémentaire d'environ 400 millions d'euros, mais je crois pouvoir dire que ces coûts sont liés, d'une part, à l'inflation des coûts énergétiques, aggravés par la guerre en Ukraine ; d'autre part, au renforcement des moyens dédiés à la cybersécurité et la quiétude de l'ordre public lors de la cérémonie d'ouverture, qui s'annonce d'ores et déjà historique. À ce jour, l'enveloppe prévisionnelle totale atteint donc 8,7 milliards d'euros.

qui connaissent une hausse de 5,8 % des crédits de paiement, soit 1,8 milliard d'euros, et une baisse de 10,8 % des autorisations d'engagement, soit 1,5 milliard d'euros. d'euros. C'est le programme 219, « Sport », dont les autorisations d'engagement sont en baisse de 22 %, qui est préoccupant pour les années à venir. Rappelons que le plan de relance complétait pour 2021 et 2022 les crédits de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » de 330 millions d'euros supplémentaires,

du sport de haut niveau, ne progressent que d'un peu plus de 2 %, ce qui est un mauvais signal à la veille de la Coupe du monde de Rugby de 2023 et des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Le dispositif Pass'Sport, soutenu de longue date par les sénateurs de notre groupe, en particulier par notre par notre rapporteur, bénéficie en 2023 d'une enveloppe de 100 millions d'euros, comme en 2022. Néanmoins, nous relevons la sous-consommation des crédits budgétaires, surprenante alors qu'il est urgent d'améliorer la condition physique dégradée de nos jeunes. Il faut donc réfléchir à une extension de l'éligibilité au Pass'Sport.

inquiétons aussi du financement du sport français, assuré pour une part importante par trois taxes parafiscales abondant l'Agence nationale du sport. Le rendement total de ces trois taxes a progressé de 9 % depuis 2017, mais la part allant au mouvement sportif a été réduite de moitié.

d'euros. Sans argent public, la volonté exprimée par le Président de la République- « Les jeux financent les jeux » -sera-t-elle respectée ? Enfin, de l'avenir du sport français à l'issue des JO ? L'examen au Sénat du projet de loi de programmation des finances publiques pour fait craindre un affaiblissement des crédits du sport après 2024. Or les JO ne doivent pas être l'arbre qui cache la forêt. Le programme 163, « Jeunesse et vie associative », bénéficie pour 2023 de 837 millions d'euros, soit une augmentation de 8,4 % par rapport à 2022.

Faut-il alors vraiment le maintenir ? Rappelons que l'objectif initial du Gouvernement était que, à l'horizon 2022, 800 000 jeunes effectuent un SNU. À titre de comparaison, le service civique, qui, lui, suscite un véritable engouement auprès de la jeunesse, ne verra ses crédits augmenter en 2023 que de 20 millions d'euros. La crise sanitaire a révélé l'importance du rôle joué par les jeunes en service civique. Alors, pourquoi ne pas renforcer encore ce dispositif, dont les crédits ne progressent que de 4 %, soit moins que l'inflation ? Un autre fait est absolument regrettable : la baisse de 10 % des crédits destinés au développement de la vie associative et au soutien du bénévolat. Très affaibli, le secteur avait déjà dû subir au début du quinquennat précédent une baisse drastique des contrats aidés, la suppression de la réserve parlementaire et, en 2020 et en 2021, la crise sanitaire. associatives redémarrent progressivement, mais les problèmes auxquels sont confrontées les associations sont encore très importants. Je le vois dans mon département du Pas-de-Calais, où les acteurs associatifs me font part de leurs difficultés, qui vont croître avec la crise économique.

Pourtant, de fortes incertitudes demeurent sur l'organisation et le financement de dispositifs absolument nécessaires à leur bon déroulement.² Pour commencer, je tiens à saluer l'esprit de responsabilité des collectivités, qui ont accepté de prendre à leur charge une grande partie des surcoûts de construction de plusieurs équipements. Pour obtenir les jeux, ses futurs organisateurs avaient pris notamment des engagements très fermes sur la réalisation d'infrastructures de transport, qui devaient permettre une circulation aisée et une consommation de carbone réduite. l'ouverture des jeux Olympiques, il faut reconnaître avec honnêteté que ces engagements ne seront définitivement pas tenus. De toutes les lignes de transport prévues dans le dossier de la candidature parisienne, une seule Il a donc été décidé de mettre en oeuvre, dans l'urgence, des transports alternatifs. Ainsi, 1 400 bus et cars spécifiques seront mobilisés, sur des voies réservées, pour les 200 000 personnes accréditées. À rebours des promesses du comité d'organisation, les jeux de Paris vont donc aggraver la pollution, accroître les embarras liés à la circulation des véhicules et dégrader davantage les conditions de déplacement des usagers des transports publics. Il est à craindre que la vie quotidienne des Franciliens ne pâtisse grandement du déroulement de ces jeux. À l'avenir, c'est l'acceptabilité de ces grandes manifestations qui est menacée. Les différents sites ont été installés à proximité de lignes que l'État, par l'entremise de la Société du Grand Paris, s'était engagé à livrer avant l'ouverture de ces jeux. Lors de son audition par notre commission, le 19 décembre 2018, M. Castex, Castex, alors délégué interministériel aux jeux Olympiques et Paralympiques, nous déclarait : « Je suis peut-être un peu " vieux jeu ", mais lorsqu'un Président de la République, un Premier ministre, quels qu'ils soient, engagent la parole de la France à l'international, spontanément, j'ai tendance à penser qu'il faut l'honorer. »

Comment cet établissement va-t-il trouver les chauffeurs nécessaires, alors qu'il en manque 1 800 en Île-de-France ? Quel est le coût de ce nouveau service et comment Île-de-France Mobilités va-t-il le financer, alors que cet organisme est proche de la cessation de paiements et que le Gouvernement et la majorité sénatoriale ont refusé, ce mercredi, de lui permettre d'accroître ses ressources financières ? Vous nous avez expliqué à plusieurs reprises, madame la ministre que les jeux devaient financer les jeux. Nous constatons aujourd'hui que ce sont les collectivités qui prennent à leur charge les surcoûts et pallient les défaillances. Les jeux ne peuvent être organisés sans argent public, mais vous avez choisi de maintenir le plafond des taxes qui financent l'Agence nationale du sport. Il est tout à fait regrettable que ce débat budgétaire ne nous ait pas permis d'apprécier plus justement les conséquences financières des manquements de l'État à ses engagements pris lors de la candidature de Paris. C'est pour cette raison que nous voterons contre les crédits

d'insertion, mais aussi de santé. La lecture du projet annuel de performance du programme « Sport » n'apaise nullement les inquiétudes que nous pouvons avoir : les crédits baisseraient de 20 % entre 2023 et 2025. Une « grande nation sportive », comme se plaît à l'évoquer le Président de la République requiert une vision budgétaire stable, claire et déclinée de telle façon qu'elle permette à l'ensemble des acteurs du monde du sport de s'engager Or ce budget, en l'état, pèche encore trop par certains aspects, notamment en dynamique de long terme et,, dans un contexte inédit d'inflation. Ainsi, au sein du programme « Sport », l'ANS bénéficie certes de 11 millions d'euros supplémentaires pour mieux structurer sa gouvernance et amplifier son action territoriale, mais les politiques publiques doivent être davantage transversales et associer

taxes dont le rendement diminue encore cette année. Il faut agir sur le plafond de ces taxes pour dégager des recettes suffisantes et financer l'ensemble des problématiques qui restent en suspens. À cet égard, nous regrettons votre obstination à ne pas vouloir que « le sport finance le sport » ! Le sport français a besoin de ressources supplémentaires pour assurer sa présence sur la durée dans tous les territoires. Nous connaissons, dans cette enceinte, le rôle massif et crucial joué par collectivités en tant que premiers financeurs publics du sport. Une nouvelle enveloppe de 100 millions d'euros est dédiée aux équipements sportifs de proximité, dans la continuité des engagements du Président de la République à « mettre le sport au coeur de la Nation », que ce soit dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques ou dans l'optique d'un enjeu d'héritage. quand on mesure l'ampleur du chantier, il semble évident qu'il manque un véritable engagement de l'État. Les collectivités ne peuvent supporter seules le coût des adaptations. On note enfin une faible progression des crédits en faveur du sport pour tous, alors que les clubs souffrent encore. Ils ont besoin de pouvoir anticiper, de se développer, de renforcer l'emploi et la formation des éducateurs et des entraîneurs pour répondre aux attentes et aux besoins des Français.

il est de bonne guerre de pointer une certaine sous-évaluation des dépenses dès le départ, conséquence d'un modèle, celui que vous nous avez présenté, dont l'équilibre était largement perfectible. Les aspects sécurité, énergie, billetterie et partenariats doivent, à terme, être maîtrisés et équilibrés, et des arbitrages doivent Comment abordez-vous cette nécessaire révision budgétaire ? Madame la ministre, il nous faut la plus grande transparence sur ces sujets, car cet événement doit rester festif et faire rayonner la France à l'échelon international. Il ne saurait se transformer en une addition douloureuse pour les Français.

Monsieur le ministre, madame la ministre, mesdames les secrétaires d'État, mes chers collègues, nous savons que l'activité physique est un outil indispensable de prévention du surpoids et de l'obésité, mais également de réussite scolaire et d'épanouissement personnel. Aussi, nous saluons les démarches du Gouvernement visant à encourager les Français, notamment la jeunesse, à prendre goût à l'activité physique, grâce à la généralisation des trente minutes quotidiennes dans toutes les écoles, l'expérimentation de deux heures supplémentaires de sport pour les collégiens et l'extension du Pass'Sport à 800 000 étudiants boursiers à la rentrée 2022. Le sport, qui permet cet épanouissement personnel physique et psychique, qui développe le goût de l'effort, de la persévérance, le respect des règles, des arbitres, des éducateurs et des adversaires, est un excellent vecteur de fraternité, nécessaire à la cohésion sociale. C'est également un excellent promoteur de l'activité physique. Aussi, je vous rappelle, madame la ministre, mon interpellation pour la promotion du sport scolaire et universitaire, qui devrait avoir une place prépondérante par rapport au « sport business » et à ses excès.

face aux restrictions d'activités, aux reports ou aux annulations de manifestations sportives et culturelles, aux résiliations d'adhésion, il proposait d'accorder un soutien financier accru aux associations. Ce texte n'a malheureusement pas été adopté. pour avis, Jacques-Bernard Magner, porte à notre attention deux éléments : la stagnation des crédits consacrés au FDVA et la complexité de certains dispositifs de soutien du tissu associatif. je prône un soutien accru à la formation dans le domaine de l'animation pour l'accueil collectif des jeunes. Madame la secrétaire d'État à la jeunesse, je vous ai interpellée ce mois-ci par une question écrite au sujet des difficultés de recrutement du secteur. L'animation n'attire plus. Certains territoires ont dû revoir à la baisse leur offre d'accueil collectif. Je proposais d'assouplir temporairement les règles d'encadrement en prévoyant un animateur pour vingt-cinq enfants par exemple, contre dix-huit actuellement, pour les enfants que l'on considère comme suffisamment je proposais d'autoriser un effectif équivalent à une classe, ce qui permettrait à de nombreuses communes de satisfaire à cette exigence. Je salue le travail fourni grâce à votre plan « Pour un renouveau de l'animation en accueils collectifs de mineurs qui dégage 5 millions d'euros d'aides pour la formation au Bafa et revalorise le contrat d'engagement éducatif. Ce cap doit être maintenu. Il faut abattre les cloisons entre l'école, la maison et la rue, agir en synergie sur les temps scolaire et périscolaire pour mieux appréhender globalement l'éducation. L'école ouverte procède de cette idée en renforçant l'articulation entre l'école et les associations, qu'elles soient sportives ou culturelles, et les communes qui les soutiennent

avec 1,1 milliard d'euros prévus pour 2023, les moyens alloués au sport restent modérés et ne représentent que 0,3 % du budget général. Cette proportion, il faut le rappeler, n'a pas évolué au cours des derniers exercices.

Ces signes sont encourageants, mais insuffisants, car une enveloppe budgétaire, même mieux dotée qu'auparavant, ne fait pas une politique. Le Gouvernement ne fait que limiter la casse et ne se donne pas les moyens de ses ambitions. Les fédérations et associations sont inquiètes : la covid-19 a fragilisé leur modèle, leurs finances, et a modifié les habitudes des usagers. Là encore, c'est au Gouvernement d'insuffler de nouveau de la confiance. Les

Or le montant des crédits alloués au renouvellement des installations locales est loin d'être à la hauteur des besoins. Et la marge de manoeuvre des collectivités, qui est limitée, ne leur permet pas toujours de maintenir en fonction certains équipements. Je pense, par exemple, aux piscines publiques, dont on connaît le rôle majeur en matière d'égalité d'accès au sport. Comment pouvons-nous afficher une priorité sur le savoir nager sans investir dans la rénovation des bassins ? appelle, une nouvelle fois, à un plan Marshall des piscines à l'échelon national, auquel seraient bien sûr associées l'ensemble des collectivités. En ce sens, une loi d'orientation et de programmation pluriannuelle du sport permettrait de mieux répondre aux enjeux des acteurs du monde associatif et des collectivités, de mieux les anticiper. Pour cela, nous avons besoin de stabilité. Nous ne voulons pas, comme cela est prévu dans le projet annuel de performance, assister à une baisse des crédits de paiement en 2024 et en 2025. Madame la ministre, quel sera l'héritage de Paris 2024 si tous les Français n'ont toujours pas accès à des installations dignes de ce nom ?

Pouvez-vous nous rassurer sur ce point, car les élus locaux comme les acteurs associatifs craignent une violente gueule de bois au lendemain des jeux ? Enfin, le Gouvernement n'a pas pris que de mauvaises décisions ; il en a aussi oublié. Je pense au sport-santé, parent pauvre de nos politiques publiques, qui ne fait l'objet que d'une action budgétaire. La promotion et le développement de l'activité physique et sportive, dans le cadre du traitement de certaines maladies, mais aussi pour notre jeunesse, apparaissent pourtant évidents. Cette mission apparaît comme une nouvelle opération de communication, dans la mesure où le Gouvernement renvoie le sport-santé à d'énièmes expérimentations, alors que l'on connaît tous ses effets positifs et que de nombreuses applications existent déjà : à Nice, à Strasbourg, à Dunkerque, à Ville-d'Avray, pour ne citer que ces villes.

Pour conclure, ce budget, qui, au premier coup d'oeil, peut sembler satisfaisant, n'est pas à la hauteur de nos ambitions. Non, le Président de la République ne peut pas décréter le sport « grande cause nationale » en 2024 et n'y consacrer que 0,3 % du budget de l'État. Mettre le sport au coeur de la Nation », c'est définir un projet ambitieux qui mobilise l'ensemble des acteurs et des territoires et prévoir les moyens budgétaires permettant de réellement répondre à tous ces enjeux. Aujourd'hui, comme notre rapporteur pour avis l'a rappelé, ces conditions ne sont pas réunies.

mais ce que je m'apprête à vous dire ne va pas forcément vous être très agréable. Je vous aime bien parce que je crois en la sincérité de votre engagement en faveur de la jeunesse pour faire de cette dernière une chance pour notre Nation. Toutefois, si je reconnais que vous êtes une croyante sincère, je regrette que vous ne soyez pas une pratiquante Nous nous retrouvons pour étudier les crédits du programme « Jeunesse et vie associative », un programme en trompe-l'oeil, comme le décrit dans son dernier rapport la Cour des comptes. Pourtant, les enjeux ne sont pas minces : la jeunesse, c'est l'avenir de notre pays, c'est notre avenir à tous.

victime d'une perte de repères sans aucun précédent. Qu'avons-nous donc à proposer à notre jeunesse ? Quelques dispositifs, mais, pour que ceux-ci forment une politique efficace, il vous manque deux choses, madame la secrétaire d'État : d'une part, une politique,

civique, laquelle dispose aujourd'hui d'une trésorerie de plus de 288 millions d'euros ! Cet argent de l'État, bien mal géré, serait plus utile à d'autres usages. On peut même parler d'un tour de passe-passe budgétaire à la Gérard Majax, référence si chère à notre Président de la République.

Votre objectif est tout autre : 64 000, soit le double des 32 000 engagés que vous avez réussi à convaincre l'année dernière, alors que votre objectif n'était pourtant que de 50 000. Là encore, c'est un tour de passe-passe budgétaire que vous nous faites, puisque, sans tenir compte des économies réalisées l'année dernière, vous promettez de budgéter les 64 000 nouveaux contrats. Ce sont donc 40 millions d'euros d'euros supplémentaires qui disparaissent. Pis encore, on s'attend d'un moment à l'autre à la généralisation de ce dispositif, qui n'a pourtant pas fait ses preuves lors de son expérimentation.

Autonomie, cohésion, service civique, sport, mixité, patriotisme, cérémonies mémorielles, rencontres, laïcité, valeurs de la République, mobilité, éducation populaire, engagement, bénévolat : quel est le point commun entre toutes ces politiques, entre

de combattre les liens de domination, de fabriquer une culture politique commune et d'en être les acteurs, en un mot de faire société en s'émancipant. Aussi, je vous propose de transférer les crédits du SNU à l'éducation populaire : nous

ont été construits au siècle passé, à une époque où l'on bâtissait vite, mais aussi- il faut le dire -assez mal. Ces équipements sportifs sont très souvent de véritables passoires énergétiques, qui font exploser la consommation d'électricité et de chauffage,

d'un tel document, ce qu'il faut, c'est de la formation et un véritable budget dédié. Il faut également créer des cellules d'écoute et d'accompagnement, auprès des clubs ou des fédérations, afin que ces pratiques se diffusent dans le milieu et que les victimes soient correctement accompagnées. Nous proposons ainsi de doubler le budget dédié à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le programme de prévention et de protection du ministère. Les bonnes intentions ne suffisent pas : elles doivent se traduire en une réelle politique.

on ne pratique pas un sport collectif en extérieur de la même manière quand il fait 25 ou 40 degrés. Au vu des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre et face à l'inaction climatique collective,

: nous proposons la création d'un observatoire de l'adaptation du sport au changement climatique afin que le Gouvernement et les autorités sportives disposent d'une instance d'expertise, d'étude et de recommandation pour la pratique sportive du futur.

Il sera surtout nécessaire de s'assurer que le déménagement du laboratoire au sein du campus Paris-Saclay, qui a pris du retard et devrait s'achever au début de l'année prochaine, se déroule dans les meilleures conditions.

de 15 à 17 ans. En outre, le présent amendement a perdu une grande part de son objet, dans la mesure où l'examen d'éventuels relèvements de plafonds de prélèvements a déjà été effectué précédemment,

S'agissant de l'amendement n° II-361, monsieur le sénateur, vous proposez de transférer quelque 14 millions d'euros alloués au SNU, afin de compenser une perte de ressources de l'Agence nationale du sport due à la baisse du rendement de la taxe Buffet.

Monsieur le sénateur Dossus, en cette Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, je ne puis que partager avec vous le constat selon lequel les violences à caractère sexiste et sexuel demeurent des fléaux dans notre société, y compris

l'enseignement de la prévention et de la lutte contre toutes les formes de violence et de discrimination dans les programmes de formation des professionnels des activités physiques et sportives. Sur le plan réglementaire également, nous allons très prochainement faire évoluer les textes régissant la préparation préparation au métier d'éducateur sportif, afin d'obliger les organismes de formation à intégrer, lors de leur demande d'habilitation, des actes de prévention de ces violences sexistes et sexuelles.

Pour assurer la mise en oeuvre des actions de formation, des financements sont accessibles aux fédérations l'Agence nationale du sport et au titre des projets sportifs fédéraux, ainsi que des projets sportifs territoriaux et des contrats de développement à national. Par ailleurs, le ministère assure le subventionnement de plusieurs associations pour des formations et des actions de sensibilisation sur cet enjeu majeur, au bénéfice des établissements sous Je n'hésiterai pas à prendre toutes les mesures qui s'imposent à l'encontre des fédérations qui ne respecteraient pas ce cadre d'action essentiel pour garantir l'intégrité du sport français.

Je tiens à souligner que la transition écologique est une priorité de tout premier plan pour mon ministère. L'adaptation de la pratique sportive au changement climatique

dernier. J'ai pu adjoindre deux volets tout à fait importants à ce plan : le déploiement accéléré de la charte des 15 engagements écoresponsables, d'une part ; l'élaboration, en lien avec le ministère de Christophe Béchu, d'un plan d'adaptation de la pratique sportive

La précédente ministre des sports avait déclaré, en février 2021, que le Gouvernement examinerait la possibilité d'augmenter la dotation budgétaire de l'ANS, en procédant au relèvement des plafonds des deux autres taxes affectées à l'Agence ou l'augmentation

Si nous voulons collectivement- le Gouvernement et le Parlement -poursuivre et véritablement renforcer le soutien aux politiques sportives, tout en préparant de la meilleure des façons l'héritage des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, alors il faudrait, comme nous l'avons plusieurs fois proposé,

La logique est simple : le sport doit financer le sport. Ces crédits supplémentaires issus des paris sportifs permettraient notamment à l'ANS de mieux flécher son soutien aux collectivités territoriales, dans le cadre du financement des équipements sportifs structurants. Nous ne voterons pas ces amendements,

Néanmoins, pour améliorer le taux de recours au dispositif, l'urgence est de renforcer les liens avec les fédérations et les associations. Il est peut-être encore un peu tôt pour modifier radicalement la gestion du Pass'Sport. La commission demande donc le retrait

le coût de la pratique peut également intégrer d'autres éléments. Le dispositif que nous vous demandons d'adopter est un message pour tous les jeunes qui veulent pratiquer le sport. Il s'agit de leur dire : « Toi aussi tu peux choisir d'avoir une activité sportive, et tu pourras la payer sans être obligé de demander à payer les 20 euros en dix mensualités de 2 euros

sein duquel les parlementaires peuvent désormais déjà siéger. Je puis témoigner de ce que j'ai vu dans la Creuse : c'est un travail sérieux. J'ai un peu moins de regrets sur la réserve parlementaire, car les fonctionnaires de l'ancienne direction départementale des sports connaissent bien le milieu associatif et font des analyses

et de la performance, parue le 22 avril 2022, quelque 84 % des sportives interrogées expliquaient vivre la période des menstruations comme une difficulté. Cet amendement vise à piloter un programme de recherche et d'actions dédié à la santé menstruelle des sportives. devra fournir des données complètes, médicales et psychologiques des sportives, mais également des préconisations pour construire des axes de formation et d'accompagnement sur mesure des sportives, des cadres et coachs, notamment les directeurs techniques nationaux et les conseillers techniques sportifs, ainsi que le recommande la boxeuse française Sarah Ourahmoune. Quel

le budget de la justice, vous me permettrez de commencer par un constat, celui qui a été dressé par le comité des États généraux de la justice : le service public de la justice est une institution qui traverse une crise majeure. C'est un bateau naufragé, qui n'a pas coulé à pic, mais qui a pris l'eau progressivement, au fil d'années de restrictions budgétaires. La crise sanitaire a, de ce point de vue, agi comme un révélateur de ses dysfonctionnements. C'est sous cet angle que nous devons analyser le budget qui nous est proposé pour l'année 2023, pour toutes les composantes de la justice : la protection judiciaire de la jeunesse, l'administration pénitentiaire, la justice judiciaire, le secrétariat général du ministère et le Conseil supérieur de la magistrature. Point positif, ce budget augmente, pour atteindre 11,6 milliards d'euros. En dix ans, les crédits alloués à la justice auront augmenté de plus de moitié. Pour ce qui concerne les effectifs, 10 000 postes devraient être créés d'ici à 2027, dont 1 500 de magistrats et 1 500 de greffiers. Les hausses successives sont absolument essentielles pour remédier aux défaillances de ce service public. Pour citer les propos de Jean-Marc Sauvé, président du comité des États généraux, « on ne peut plus continuer d'appliquer une multitude de rustines à une chambre à air dont on n'a pas voulu voir qu'elle était totalement usée. » Une réforme systémique s'impose, tant sur le fond que sur le plan du budget. Monsieur le ministre, la future loi de programmation qui, je l'espère, nous sera prochainement présentée devra consacrer cette trajectoire. Il ne s'agira bien sûr pas de vous donner un blanc-seing ! L'augmentation significative des moyens du ministère de la justice depuis plusieurs années doit s'accompagner de la diffusion d'une réelle culture de l'évaluation des dépenses réalisées. Telle que je la conçois, une loi de programmation ne doit pas simplement consister en la définition d'indicateurs de performance et de lignes de crédits et d'emplois. Elle doit être l'occasion, pour le ministère concerné, de s'interroger sur le sens des politiques publiques qu'il mène, sur la qualité du service public qu'il soutient et sur sa propre gestion des moyens, budgétaires comme humains. la future loi de programmation des moyens de la justice ne pourra faire l'économie d'une réflexion sur l'amélioration de la gestion et sur la construction d'indicateurs de suivi fiables. Le ministère s'est trop longtemps retrouvé « dans l'incapacité de relever les défis d'une gestion rigoureuse », pour reprendre de nouveau un constat des États généraux. Prenons l'exemple du plan de transformation numérique de la justice (PTN), initialement doté de 530 millions d'euros. Il est inconcevable que, comme elle l'a admis dans un rapport remis à la demande de la commission des finances, la Cour des comptes ait rencontré d'importantes difficultés pour reconstituer les dépenses budgétaires exécutées au titre du PTN L'informatique fait d'ailleurs partie, avec l'immobilier et la gestion des ressources humaines, des trois chantiers qui doivent être menés à bien pour soutenir le service public de la justice. Je suis en effet convaincu que l'institution judiciaire ne sortira pas de sa crise majeure si elle ne s'interroge pas sur la gestion de ses fonctions support, faut rapprocher des utilisateurs, avec un impératif : mieux prendre en compte les besoins des usagers de la justice, qu'il s'agisse des personnels, des justiciables ou des professionnels du droit, tels que les avocats. l'informatique, un second plan de transformation numérique est amené à prendre la suite du premier, établi pour la période 2018-2022. La commission des finances avait entendu la Cour des comptes sur sa mise en oeuvre au mois de février dernier. Soyons clairs : si le premier plan de transformation numérique était un plan de rattrapage, le second devrait être celui de la modernisation. Pour réussir, il devra non seulement être doté de moyens budgétaires suffisants, mais également tenir compte de plusieurs impératifs. Il devra tout d'abord pleinement inclure les usagers et leurs besoins, alors que le malaise grandit au sein des juridictions sur les outils numériques. Il n'est pas normal que la modification de certains systèmes d'information oblige désormais les magistrats et les greffiers à ressaisir manuellement certaines données Ensuite, le second PTN devra conduire à une véritable interopérabilité des systèmes d'information du ministère. Par exemple, aucune application ne permet aujourd'hui de fournir des données sur le parcours complet complet des mineurs pris en charge par la justice. Le décloisonnement des applications devra donc s'opérer en interne, mais aussi en externe, avec le ministère de l'intérieur par exemple, ainsi qu'avec les professionnels du droit, comme les avocats. Le deuxième enjeu est celui de la professionnalisation de la gestion des ressources humaines. Je suis convaincu que le pilotage des ressources humaines n'est pas seulement une question d'augmentation des effectifs : il implique également de prendre en compte les questions relatives au vivier de recrutement au vivier de recrutement ou à la revalorisation de certains métiers en perte d'attractivité. Il s'agit là d'un enjeu capital, qui ne peut se contenter d'une seule réflexion sur la rémunération. J'en viens à la troisième fonction support : l'immobilier. Le plus grand chantier du ministère est, bien sûr, celui de la construction de 15 000 places de détention supplémentaires, sous l'égide de l'administration pénitentiaire. Je reste toutefois persuadé- nous aurons l'occasion de vous entendre à ce sujet, monsieur le garde des sceaux, lors de la discussion de l'article 44 -qu'une politique pénitentiaire ne peut se résumer à une politique immobilière. À l'inverse, la politique immobilière du ministère ne peut se résumer au « plan 15 000 ». Les programmes de rénovation, que ce soit des tribunaux judiciaires ou des établissements de détention, sont absolument cruciaux. Ils participent aussi de la valorisation des magistrats, des greffiers ou des surveillants pénitentiaires. Au regard des missions absolument essentielles que ceux-ci accomplissent, nous leur devons d'améliorer leurs conditions d'exercice. Telles sont, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, les observations que je souhaitais formuler sur le projet de budget du ministère de la justice.

avis. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, pour la troisième année consécutive, les crédits alloués à l'administration pénitentiaire dans le projet de loi de finances s'inscrivent en forte hausse, avec une progression de 7,5 %. Ces moyens supplémentaires ne sont pas superflus, compte tenu des besoins en moyens humains et des investissements nécessaires pour rénover et développer notre parc pénitentiaire. Pourtant, les auditions auxquelles j'ai procédé m'ont parfois donné l'impression que les efforts réalisés sur le plan budgétaire n'avaient pas encore d'effets perceptibles sur le terrain. Je vois à cela deux explications : tout d'abord, une part importante des crédits est absorbée par le « programme 15 000 », qui vise à ouvrir 15 000 nouvelles places de prison d'ici à 2027 ; ensuite, le retour à une situation de surpopulation carcérale dégrade les conditions de travail du personnel, ainsi que les conditions de détention. Concernant le « programme 15 000 », je rappelle qu'il est divisé en deux tranches : 7 000 places devaient être livrées entre 2017 et 2022, et 8 000 entre 2022 et 2027. Nous devons constater que la première tranche a pris du retard, puisque le nombre de places livrées en cette fin d'année 2022 est de l'ordre de 2 000. La livraison d'une dizaine d'établissements est prévue en 2023, ce qui permettra de combler une partie de ce retard. Il n'en reste pas moins que l'achèvement du programme à l'échéance prévue paraît aujourd'hui bien incertain. Je m'interroge, en particulier, sur les surcoûts qui résulteront de la hausse des prix de l'énergie et des matières premières : ils pourraient inciter à étaler dans le temps la mise en oeuvre du programme. Après la baisse constatée en 2020, du fait de la pandémie, la population carcérale est repartie à la hausse, pour se rapprocher désormais de ses plus hauts niveaux historiques. Dans les maisons d'arrêt, le taux d'occupation dépasse 140 % en moyenne, avec des pointes à plus de 200 % dans certains établissements, par exemple à la prison de Bordeaux-Gradignan, sur laquelle la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté nous a alertés. Dans ce contexte, le Gouvernement a fait adopter, à l'Assemblée nationale, un amendement tendant à reporter une nouvelle fois la mise en application du principe de l'encellulement individuel. À l'évidence, les conditions observées sur le terrain font obstacle au respect de ce principe à compter du 1 janvier 2023. La surpopulation carcérale dégrade tout d'abord les conditions de détention on observe davantage de matelas au sol et un accès plus difficile aux activités sportives ou culturelles, et le suivi par les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation (CPIP) tend à s'espacer, ce qui réduit les chances de réinsertion. Elle détériore également les conditions de travail du personnel les schémas d'emplois dans les établissements sont définis en fonction du nombre théorique de places, non en fonction du nombre de détenus réellement accueillis ; d'où une importante surcharge de travail, notamment pour les surveillants pénitentiaires, qui sont quotidiennement au contact des personnes incarcérées. En dépit de ces difficultés qui persistent, la commission des lois a émis un avis favorable sur l'adoption des crédits de l'administration pénitentiaire, ainsi que sur l'article rattaché 44 , tout en étant convaincue de la nécessité de remettre à niveau de notre service public pénitentiaire.

généraux de la justice, ils sont toujours dans la rue. Or le projet de budget pour 2023 poursuit l'effort de rattrapage, avec une hausse des crédits de paiement de 8 %, dont 300 millions d'euros supplémentaires pour les juridictions. les juridictions. Pourquoi, alors que le budget de la justice augmente pour la troisième année consécutive, le malaise persiste-t-il ? Pourquoi, malgré les recrutements en nombre, les délais de jugement s'allongent-ils toujours, passant, pour les affaires civiles, de 11,4 mois en 2019 à 13,7 mois en 2021 et à près de 50 mois pour les crimes ? La création, en 2023, de 1 220 postes, dont 546 titulaires- 200 magistrats, 191 greffiers et 155 directeurs de greffe doit permettre de renforcer les juridictions. Cette dynamique devrait se poursuivre avec la création, sur cinq ans, de 1 500 postes de magistrats, 1 500 postes de greffiers et 2 000 postes de juristes assistants. Ces moyens humains sont

les moyens de formation des personnels recrutés et d'attirer de nouvelles vocations. Pour cela, le PLF prévoit une prime de 1 000 euros brut en moyenne pour les magistrats judiciaires, modulée en fonction de l'ancienneté. Pour les greffes, un effort de 165 euros brut par mois pour les greffiers et de 250 euros pour les directeurs de greffe est prévu. Cette augmentation est la reconnaissance du rôle central des greffiers dans la chaîne judiciaire, mais elle ne permettra pas l'amélioration réelle de leurs conditions de travail tant qu'il y aura 7 % de postes non pourvus et que les conditions matérielles- informatiques et locaux -ne seront pas améliorées. Je pense particulièrement au greffe du tribunal judiciaire de Rouen, qui travaille dans des conditions peu acceptables : pas de fenêtres, bureaux partagés avec la salle de pause des agents ou installés dans d'anciennes toilettes réaffectées, faute de place. Cependant, cette augmentation massive des effectifs doit impérativement s'accompagner d'une véritable politique de ressources humaines. L'évaluation de la charge des magistrats, que nous appelons de nos voeux depuis cinq ans, devrait heureusement aboutir à la Mais il importe surtout de moderniser les méthodes de travail du magistrat, en créant une « équipe », qui lui permettra de se concentrer sur son office, de revaloriser le rôle des greffiers et de donner un avenir aux contractuels. Cela nécessitera une clarification des missions de chacun, aujourd'hui peu lisibles, entre les assistants de justice, les juristes assistants, les contractuels « justice de proximité » et les assistants spécialisés sceaux, vous vous êtes engagé sur le chemin long et sinueux de la réforme de la justice. Si nous considérons qu'il faut aller plus vite, il convient surtout d'éclaircir la méthode ! Les États généraux de la justice donnent le guide ; il faut maintenant fixer le cap. Ce budget est un bon début. C'est pourquoi la commission des lois a émis un avis favorable. La parole est

augmentent encore une fois, certes. Pourtant, force est de constater que, sur le terrain, en dehors de l'aspect matériel, les évolutions concrètes sont encore attendues. Nous le signalons chaque fois que nous en avons l'occasion, depuis plusieurs années maintenant, et nous continuerons à le faire. D'ailleurs, si j'en crois, « après le naufrage de la numérisation des procédures civiles pilotée par Sopra Steria et Cap Gemini, le ministère a signé un nouveau marché de 45 millions d'euros

Parlons des victimes de violences conjugales, qui représentent plus de 40 % des personnes prises en charge par les associations d'aide aux victimes. Le budget pour 2023 permettra de financer 5 000 téléphones grave danger et 835

? Malheureusement, même lorsque la victime a la chance d'être reconnue par l'institution, elle se heurte trop souvent à de grandes difficultés dans le traitement de son dossier, voire de ses dossiers-

concrètes sur ce sujet. Je puis d'ores et déjà vous dire que les trois premières d'entre elles seront : formations, formations et formations ... En effet, on ne peut pas traiter correctement ces dossiers si l'on ne sait pas ce que sont le psychotraumatisme, l'emprise ou encore le contrôle coercitif, et ce que cela entraîne chez la victime. Aussi, je vous remercie de cette mission et, même si

Dans le prolongement des années précédentes, je souhaite me concentrer sur trois défis majeurs auxquels fait face la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) : la redynamisation du milieu ouvert, les difficultés de recrutement et la mise en oeuvre progressive de l'applicatif métier Parcours. Le code de la justice pénale des mineurs (CJPM) est en vigueur depuis maintenant un peu plus d'un an. Nous savons qu'il a entraîné un bouleversement de la manière de travailler des services placés auprès des juridictions, dont l'activité a considérablement augmenté, d'après les premiers retours sur la réforme. Toutefois, cette réforme a aussi et peut-être surtout un impact sur le milieu ouvert, soumis à la nécessité d'organiser une prise en charge avant l'audience de sanction. Le CJPM peut être un levier de la redynamisation du secteur ouvert ; c'est l'un des axes de travail de la PJJ, qui s'appuie sur les Assises du placement judiciaire, closes en octobre dernier. L'attention croissante portée au milieu ouvert, notamment par des créations de postes et les moyens donnés aux unités éducatives d'accueil de jour, est bienvenue. Au cours des dernières années, nous avons en effet eu l'occasion de nous inquiéter de la place très importante prise par la création des centres éducatifs fermés (CEF) dans l'augmentation du budget de la PJJ- elle en a représenté près d'un quart sur les trois dernières années -, alors même que les besoins du milieu ouvert sont très importants. J'en viens justement à la question des centres éducatifs fermés, dont le développement a constitué un axe majeur de la politique du Gouvernement ces dernières années. Sur le programme de 20 nouveaux CEF, il semble aujourd'hui que la PJJ soit amenée à renoncer à trois ou quatre projets, qui ne pourront aboutir. Parallèlement, deux nouveaux projets de CEF sont envisagés. Sous-jacente aux difficultés de la PJJ est la question des personnels. Il s'agit là d'une véritable inquiétude, en raison d'un taux de vacance de postes de 6 % et d'un niveau de rotation élevé sur plusieurs postes difficiles. Le taux de contractuels dans la PJJ, supérieur à 20 %, et celui de leur renouvellement sont eux aussi élevés. Si de nouveaux postes sont créés chaque année, nous avons noté, par le passé, que tous ne parviennent pas à être pourvus. Face à ce manque d'attractivité, la revalorisation salariale est nécessaire, mais elle n'est apparemment pas suffisante, au moins à court terme. Il faut également redonner du sens aux métiers de la PJJ, avec des orientations mobilisatrices et la volonté d'agir pour l'insertion des jeunes. Les moyens déployés à cette fin peuvent aller en ce sens. Je veux, pour terminer, évoquer le déploiement de l'applicatif Parcours. L'appropriation de l'outil s'est révélée particulièrement difficile, et le besoin de formation est important. La PJJ a donc relancé un programme de formation des personnels. De nouveaux développements se révèlent nécessaires, mobilisant 4 millions d'euros en 2022 et, de nouveau, en 2023, pour permettre le déploiement du deuxième lot de Parcours, destiné aux éducateurs eux-mêmes. Pour l'heure, au regard de l'augmentation de son budget, la commission des lois a émis un avis favorable sur l'adoption des crédits du programme 182. Mes chers 182. Mes chers collègues, je vous rappelle que le temps de parole attribué à chaque groupe pour chaque discussion comprend le temps de l'intervention générale et celui de l'explication de vote. Par ailleurs, le Gouvernement dispose au total de quinze minutes

Certes, ces États généraux ont permis de renouer un dialogue perdu entre les acteurs de la justice et les pouvoirs publics. Le budget, sur les trois dernières années, bénéficie d'une augmentation significative de ses crédits. Nous devrions nous féliciter de cette prise de conscience, mais, derrière les effets d'annonces, la réalité est hélas plus compliquée. Les difficultés structurelles des juridictions sont considérables, et notre système judiciaire est à bout de souffle. La justice française est l'une des plus mauvaises élèves de l'Union européenne. Elle compte trois procureurs pour 100 000 habitants, contre 12 en moyenne dans les États membres. Son budget demeure inférieur à celui des autres pays européens comparables. Avec un budget de 5 euros par habitant consacré à l'aide juridictionnelle, la France se situe encore en dessous de la moyenne européenne, qui est de 6,50 euros par habitant. Un exemple très parlant illustre les défaillances et l'encombrement de notre justice : une dépêche interministérielle, datée de mai 2021, a incité les magistrats à classer sans suite de très nombreuses affaires jugées trop anciennes ou pour lesquelles aucune enquête n'a été menée. Ces injonctions illustrent tout l'échec de notre système judiciaire. La justice française souffre également d'une sous-évaluation chronique des besoins humains dans les juridictions. À titre d'exemple, le taux de vacance des postes de greffier s'établit à 7,2 %, soit 2,7 points de plus qu'en 2019, avant la crise du covid-19. Les embauches de près de 200 magistrats et 198 greffiers ne pourront, hélas, répondre aux besoins que représentent les postes non pourvus. Sur ces postes, nous dénonçons également la méthode du Gouvernement consistant en une embauche massive de contractuels. Ces assistants de justice contractuels, en situation précaire, remplacent à bas coût les recrutements de magistrats. Cette politique de recrutement à moindre coût n'est pas une solution pérenne acceptable pour notre pays, la logique gestionnaire à courte vue qui s'impose de plus en plus, au détriment de la qualité de la justice rendue et de l'accès à la justice pour tous les citoyens. Des moyens supplémentaires seront, en outre, alloués au bracelet anti-rapprochement. Or ces outils, dès leur création, ont connu de nombreux dysfonctionnements techniques, ce qui a conduit le ministère à changer de prestataire en 2022. Cet exemple montre que, en dépit de moyens supplémentaires, le pilotage fait toujours défaut Enfin, que dire du budget colossal alloué à la construction de nouvelles prisons ? En dépit des nombreuses condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) pour les conditions indignes de détention, aucune réflexion n'est menée sur l'architecture des parcs actuels et sur l'entretien des établissements existants, alors que cela permettrait d'améliorer rapidement la qualité de vie des détenus et les conditions de travail des surveillants pénitentiaires. La promesse des 15 000 places pour 2027, défendue comme remède aux problèmes chroniques de surpopulation, nous paraît inappropriée. Le taux d'occupation des places en maison d'arrêt pourrait ainsi atteindre plus de 130 % en 2023. Les subventions aux associations, destinées à financer les activités culturelles et sportives des détenus, connaissent une diminution importante, de 25 %, alors que les activités organisées au sein de la détention participent au quotidien carcéral et s'inscrivent pleinement dans le parcours de réinsertion. Dans ces conditions, comment espérer une véritable amélioration des conditions de détention ? des sceaux, des créations de postes de surveillant, mais nous savons tous ici que ce budget sera difficile à mobiliser, puisque cette profession souffre, en vérité, d'une grave crise des vocations, en raison notamment des conditions de travail et de rémunération, qui ne sont pas à la hauteur des enjeux et des missions effectuées par ces agents. mots porteront sur la protection judiciaire de la jeunesse, qui, au gré des réformes et des budgets, reste le parent pauvre de la justice. Certes, la PJJ bénéficie d'une hausse budgétaire, mais la priorité donnée par le Gouvernement est fléchée vers la création de places dans les centres éducatifs fermés ou renforcés. La culture du tout-répressif a ses limites, surtout pour ce qui est de notre jeunesse, même lorsqu'elle est délinquante. C'est pourquoi, même si, dans son ensemble, nous saluons l'augmentation du budget de la mission « Justice », la répartition des crédits ne répond pas suffisamment aux besoins de recrutement de personnels, aux difficultés de la justice du quotidien ni au besoin d'améliorer rapidement les conditions de détention dans notre pays. Notre groupe s'abstiendra donc sur les crédits de cette mission. La parole

un budget important pour 2023, puisque les crédits alloués au ministère de la justice augmentent de nouveau de 8 %. Cette hausse est d'autant plus opportune que les États généraux de la justice ont mis en exergue l'impérieuse nécessité de maintenir une trajectoire ambitieuse. Cela a été rappelé à de nombreuses reprises : le budget de la justice a augmenté de 26 % depuis votre entrée au Gouvernement et de 40 % depuis le début du premier quinquennat du président Macron, ce qui est considérable. Certes, notre enthousiasme doit être tempéré, car ce changement de braquet, opéré depuis trois ans, n'inverse pas encore la tendance. La France demeure l'un des pays d'Europe qui consacre le moins d'argent à sa justice.

Cependant, nous ne serions pas honnêtes si nous ne reconnaissions pas les grandes avancées que permettra ce beau budget. Je pense tout d'abord aux moyens humains, puisque ces crédits rendront possibles un renforcement des effectifs- 2 253 emplois seront créés cette année -, ainsi que l'amélioration des conditions de travail des agents et de la qualité du service rendu. Ainsi, 80 millions d'euros sont prévus pour revaloriser les salaires de tous les agents du ministère, des magistrats, qui verront leur rémunération augmenter de 1 000 euros bruts par mois en moyenne, jusqu'aux éducateurs, en passant par les surveillants pénitentiaires. Le budget permettra également de poursuivre les programmes immobiliers judiciaires et pénitentiaires. S'agissant de l'administration pénitentiaire, et alors que nous connaissons un retour à une surpopulation carcérale endémique, le Gouvernement a décidé de poursuivre la sécurisation et la modernisation du service public pénitentiaire. La création de nouvelles places de prison dans le cadre du « plan 15 000 » doit nécessairement s'accompagner du développement des aménagements de peines et des mesures alternatives à l'incarcération. À ce titre, je salue les efforts déployés par le Gouvernement pour favoriser la réinsertion des personnes placées sous main de justice et me réjouis de la hausse des crédits consacrés à la mise en place du statut du détenu travailleur, qui aidera à prévenir la récidive et à maintenir un climat apaisé en détention. La hausse des moyens consacrés au renforcement de la sécurité des personnels et des établissements est à souligner également. La montée en puissance du rôle du surveillant pénitentiaire, l'ouverture de nouvelles unités pour détenus violents, la généralisation des caméras-piétons sont autant de mesures qui permettront de lutter plus efficacement contre les violences au sein de nos établissements pénitentiaires. Enfin, des efforts renouvelés et importants sont déployés en faveur de la modernisation de la justice et du renforcement de l'accès au droit. Aussi, je souhaite souligner l'augmentation des crédits destinés aux investissements numériques, des crédits consacrés aux frais de justice pour renforcer notamment les moyens d'enquête et d'expertise judiciaire, des crédits dédiés à l'accès au droit et à la médiation, des crédits alloués à l'aide juridictionnelle, ou encore des crédits affectés à l'aide aux victimes- à l'aide aux victimes- cette hausse contribuera à une meilleure justice de proximité. Monsieur le garde des sceaux, je manquerais à tous mes devoirs si je ne vous réinterrogeais pas sur les annonces que vous avez faites lors de votre déplacement à Mayotte en mars dernier. Je pense particulièrement à la création d'une nouvelle cité judiciaire, d'un second centre pénitentiaire ou encore d'un centre éducatif fermé. Comprenez mon insistance, mais j'espère que vous pourrez nous apporter de nouvelles précisions sur leur calendrier de mise en oeuvre. La réalisation de ces projets prendra nécessairement du temps, d'autant que nous faisons face à un énorme problème de foncier, lequel pourrait retarder la concrétisation de ces indispensables évolutions. que peut-on entreprendre immédiatement pour traiter et juguler la terrifiante flambée de la délinquance juvénile que l'on peut observer sur place ? Le groupe RDPI, que je représente, considère que ce budget dote le ministère de la justice de moyens à la hauteur de ses missions, car il accélérera sa modernisation et mettra en oeuvre les recommandations issues des États généraux de la justice, ainsi que les mesures contenues dans la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire.

allons-nous saluer l'augmentation de 7,8 % des crédits de la justice, soit 710 millions

garde des sceaux, que vous aurez à coeur de prendre en compte les conclusions de ce travail accompli par le Sénat. En ce qui concerne l'administration pénitentiaire,

et dorment sur des matelas au sol, au mépris de toutes les conditions d'intimité que l'on est en droit d'attendre dans nos prisons.

pour combler les difficultés structurelles de la justice, car nous partons de trop loin. L'institution judiciaire est dans un état plus que dégradé, et les crises internes qu'elle subit exigent que nous agissions en responsabilité.

Face à cela, vous concentrez les moyens sur l'extension du parc carcéral, une mesure qui, de surcroît, ne permettra pas de résoudre le problème de la surpopulation. À ce À ce propos, rappelons que les taux d'incarcération et de surpopulation carcérale en France sont parmi les plus élevés d'Europe. Les conditions de détention indignes dans les prisons françaises sont régulièrement dénoncées depuis de nombreuses années,

ses personnels sont souvent en souffrance et démotivés. Parmi les annonces récentes, l'augmentation de traitement substantielle dont vont bénéficier les magistrats en 2023 est naturellement une très bonne chose. Elle leur permettra d'être rétribués,

il en faut pour les personnels de votre ministère ! Il en faut aux surveillants pénitentiaires, qui souffrent d'un déficit d'image ; il en faut aux greffiers, ainsi qu'aux magistrats traitant de la justice pénale. J'entendais encore cette semaine, à l'occasion d'un rassemblement devant le

pourtant tous ici que, en vertu du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue [ ...] dans un délai raisonnable, par un tribunal ». Lors d'un récent déplacement au Québec,

Nous aurons l'occasion d'aborder de nouveau ces sujets dans le cadre du projet de loi de programmation qui est encore en préparation et qui prendra la suite de la loi portée par votre prédécesseur pour la période 2018-2022. Ce texte nous permettra, au-delà de la discussion budgétaire 2023, d'aborder la question des investissements à long terme de votre ministère, notamment en matière immobilière. Comme vous l'avez rappelé lors de votre audition devant notre commission, il faut prévoir et préparer l'accueil des recrutements que vous avez annoncés. Cela passe par des investissements massifs dans l'immobilier de nos juridictions, qui en ont cruellement besoin. Il convient de mieux accueillir les justiciables, bien sûr, mais aussi d'améliorer les conditions de travail des agents actuels et des renforts humains qui les rejoindront au cours des cinq années à venir. En la matière, la marge de progression est importante. On peut regretter, au-delà de l'état général de certains bâtiments, le manque d'autonomie dans la gestion du quotidien des tribunaux. des tribunaux. Remplacer une ampoule, effectuer des travaux d'entretien ou des réparations basiques : autant de tâches pour lesquelles chaque chef de juridiction devrait être capable d'agir rapidement et de manière autonome,

Avec un taux d'encellulement individuel de seulement 20,1 %, il était, certes, illusoire de penser que nous serions capables de respecter ce principe au 31 décembre 2022. Pour autant, nous ne cessons de prolonger ce moratoire depuis la loi pénitentiaire de 2009,

Monsieur le garde des sceaux, nous saluons les arbitrages budgétaires que vous avez réussi à obtenir dans le cadre de la mission « Justice » du PLF pour 2023. Le groupe Union Centriste apportera donc son soutien à ses crédits, et nous attendons avec impatience et vigilance de loi de programmation, en espérant que celui-ci permettra d'inscrire dans la durée le rattrapage du retard accumulé ces dernières décennies. Gardons à l'esprit que la France consacre aujourd'hui 72,50 euros par habitant à son système judiciaire, près de deux fois moins que l'Allemagne, et qu'elle est le seul des grands pays européens à dédier moins de 0,3 % de son PIB à la justice.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mesdames, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord évoquer la mémoire de Charlotte, l'histoire tragique d'une jeune magistrate de 29 ans qui s'est donné la mort le 23 août 2021 à Béthune. Envoyée de tribunal en tribunal, elle comblait les effectifs manquants des juridictions du Nord. À ces conditions de travail difficiles s'ajoutaient des injonctions à aller toujours plus vite, symptôme d'une justice malade qui préfère un jugement rapide et dégradé à un jugement de qualité. À la suite de son suicide, une pétition réunissant 3 000 magistrats et plus de 100 greffiers a vu le jour pour condamner une justice qui n'écoute pas et qui chronomètre tout. Parlons de la magistrate Marie Truchet, qui s'est écroulée en pleine audience de comparution immédiate, le 18 octobre dernier, au tribunal de Nanterre, pour ne plus jamais se relever.

une illustration supplémentaire du ras-le-bol qui règne au sein du corps judiciaire. Dans son rapport, le comité des États généraux met également l'accent sur l'importance de la réinsertion en prison. une augmentation significative des crédits alloués à l'insertion professionnelle des détenus, dont 2,8 millions d'euros pour le renforcement du statut de détenu travailleur et 2 millions d'euros consacrés à la diversification des actions de réinsertion. J'aurais aimé que l'on s'indigne autant de l'état de nos prisons que d'une séance de karting à la maison d'arrêt de Fresnes ... Mes nombreuses visites en prison me permettent d'attester que les prisons françaises ne répondent pas à l'exigence de dignité tout être humain peut prétendre. Nous ne soignerons pas le fléau de la surpopulation carcérale par l'élargissement du parc immobilier. La solution est ailleurs

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mesdames, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, voilà maintenant trois ans que la justice de notre pays rattrape progressivement son retard budgétaire. Nous partions de très

de ce budget : financement des revalorisations indemnitaires des magistrats et des greffiers ; mise en oeuvre des recrutements nécessaires ; nouvelle hausse des crédits budgétaires portée par l'augmentation des frais de justice et par l'immobilier judiciaire ; développement des aménagements de peines et des mesures alternatives à l'incarcération. Tout cela nous semble aller dans la bonne direction. Pour 2023, les crédits de la mission « Justice » connaissent une augmentation inscrite dans la continuité des deux exercices budgétaires précédents, et la dynamique observée en matière d'emplois doit être soulignée. J'y insiste, tant les maux de la justice dans notre société se résument souvent à des questions de temps. D'un côté, le temps d'attente d'un jugement est trop long pour le justiciable, dont l'impatience se justifie ; de l'autre, le temps disponible pour les juridictions est trop limité, ce qui entrave leur capacité à rendre des décisions suffisamment motivées et comprises par nos concitoyens.

Tout le monde pense spontanément à la justice pénale, mais d'autres services sont également sinistrés. J'ai en particulier à l'esprit la protection judiciaire de la jeunesse. De nombreux établissements qui en relèvent sont saturés en raison d'un manque de personnel et font face à des difficultés de recrutement, comme l'a souligné notre collègue Maryse Carrère,

sa complexité permet de garantir que les décisions qui en émanent sont équilibrées et répondent aux vertus de prudence, de tempérance, de justice et de force auxquelles notre République aspire. Aussi, à des procédures simplifiées, nous préférons un renforcement des moyens, humains comme matériels, et des formations. Les magistrats, greffiers et avocats expriment régulièrement leur mal-être, par des grèves ou des tribunes de presse ils nous font part de leur surcharge de travail, de leur découragement et de leur épuisement. Je suis certain, toutefois, qu'aucun d'entre eux ne voudrait renoncer aux principes fondamentaux de notre justice. Nous devons donc continuer à former et à recruter, sans jamais dévoyer notre droit processuel. Pour ce faire, il faut des moyens. Ce budget en comporte, nous le saluons, mais l'effort n'est pas encore achevé. Le projet de loi de programmation qui est annoncé devra s'inscrire dans cette dynamique. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, tout en restant vigilant, le groupe du RDSE votera en faveur des crédits de cette mission.

se traduisant par un projet de loi de programmation pour la justice, élaboré dans une grande concertation et fondé sur une étude d'impact approfondie, soumise au Parlement.

au point que les conditions d'exercice des professionnels du droit sont devenues insoutenables. Au point, aussi, que nos concitoyens ont perdu confiance en elle : en juillet dernier, 70 % des Français considéraient que la justice fonctionnait mal. Lorsque l'on sait le rôle essentiel que cette institution joue dans notre société, aussi bien pour la cohésion nationale que pour la vie de notre démocratie, nous ne pouvions que nous en inquiéter. Il était urgent d'inverser la tendance. Le budget de la justice progresse ainsi de 26 % entre 2020 et 2023. Comme la commission, nous notons la place prépondérante de l'administration pénitentiaire dans ce budget. La construction de places de prison est une nécessité pour assurer le respect de notre politique pénale. pénale. Elle s'impose aussi pour éliminer la surpopulation carcérale et permettre à notre pays de respecter ses engagements en matière de droits humains. Les juridictions judiciaires ont également un impérieux besoin de crédits. Les magistrats sont débordés, et ils sont depuis longtemps en nombre insuffisant.

Autre mesure très attendue de ce projet de budget, les magistrats judiciaires vont bénéficier d'une revalorisation indemnitaire de 1 000 euros brut. Cette revalorisation nous paraît nécessaire pour maintenir l'attractivité de la fonction. Elle contribuera également à mettre fin à une inégalité entre les magistrats judiciaires et les magistrats administratifs ou financiers qui ne se justifiait nullement et à laquelle il est grand temps de mettre un terme.

Ce n'est pas à vous, monsieur le garde des sceaux, que nous apprendrons le rôle essentiel des avocats. Auxiliaires de justice, ils assurent la défense de nos concitoyens et se battent pour faire respecter leurs droits et libertés. Cette mission est encore plus nécessaire auprès de ceux de nos concitoyens qui sont les plus démunis. Le budget de cette année prolonge la dynamique de l'augmentation de la rétribution des avocats d'aide juridictionnelle. Il s'agit ici non pas d'intérêts catégoriels, mais bien de l'accès au droit et au juge. Nous nous félicitons donc de cette augmentation. Le volet numérique qu'évoquait François-Noël Buffet constitue aussi un chantier important. Comme beaucoup d'autres, le ministère de la justice fait face à des difficultés dans la numérisation de ses activités. Nous souhaitons tous que l'augmentation du budget de la justice produise ses effets le plus rapidement possible. Les délais de jugement sont encore beaucoup trop longs : plus d'un an pour une affaire civile, deux ans pour un divorce et plus de quatre ans pour une affaire pénale. Nous ne pouvons pas nous en satisfaire. La justice prend du temps, mais tant qu'elle n'est pas passée, l'application du droit est comme suspendue. Les augmentations de budget comme celles de ces dernières années contribuent à améliorer la justice de notre pays et à renouer la confiance entre les citoyens

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mesdames, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues,

le comité des États généraux de la justice avait affirmé dans son rapport le besoin de ce rehaussement budgétaire, mais il précisait aussi la nécessité de repenser de façon systémique et articulée l'institution judiciaire, en soulignant que, avant de poser la question des moyens, il fallait clarifier les objectifs assignés à la justice.

le projet de budget que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui devrait permettre, si vous le votez, une nouvelle hausse de plus de 8 % en 2023 au profit de notre justice. sont ainsi 710 millions d'euros supplémentaires qui abonderont en 2023 le budget du service public de la justice, qui frôlerait ainsi les 10 milliards d'euros pour l'année 2023. D'aucuns diront peut-être que ce n'est toujours

en 2023, soit une hausse de plus de 26 % du budget en trois ans, et de plus de 40 % si l'on prend comme point de départ le début du premier quinquennat du Président de la République. Pour mémoire, le budget de la justice s'élevait, en 2017, à 6,9 milliards d'euros. Cette nouvelle hausse budgétaire confirme la priorité pluriannuelle donnée à la justice au sein de la politique gouvernementale. Elle confirme notre cap : continuer le rattrapage de trente ans d'abandon de la justice et mettre en oeuvre les recommandations issues des États généraux de la justice.

des emplois en juridiction, dont 605 ont d'ores et déjà été pérennisés au titre de la justice de proximité à la mi-2022. Ces 10 000 recrutements seront répartis finement, année après année, en fonction des besoins qui nous remontent du terrain, mais également des besoins opérationnels. opérationnels. J'ai toutefois sanctuarisé la création de 1 500 postes de magistrats et de 1 500 postes de greffiers supplémentaires sur tout le quinquennat, afin de renforcer les effectifs en juridiction.

Ces 2 253 personnels seront répartis de la façon suivante : 1 220 pour la justice judiciaire, dont 200 magistrats et 191 greffiers,

en sus de ces 2 253 emplois supplémentaires, 60 sont prévus pour nos opérateurs. Deuxièmement, mesdames, messieurs les sénateurs, pour assurer ce niveau inédit de recrutement, je souhaite renforcer encore l'attractivité des métiers de la justice par des revalorisations salariales. À cet effet, le budget 2023 permettra, une fois encore, d'augmenter les crédits alloués au titre des mesures catégorielles,

Concernant les personnels relevant des corps spécifiques de la protection judiciaire de la jeunesse, 7 millions d'euros seront consacrés cette année à des revalorisations indemnitaires. Nous achevons en

Les surveillants pénitentiaires ont de plus bénéficié en 2022 d'une réforme importante de leur statut et de leur rémunération. La fusion des grades de surveillant et de et de brigadier a permis de simplifier la carrière des agents et de revaloriser les rémunérations, notamment en début et en fin de carrière.

ces crédits permettront au ministère d'achever le plan de construction des 15 000 places de prison supplémentaires voulu par le Président de la République. Ce plan permettra d'augmenter la capacité carcérale de 60 000 à plus de 75 000 places.

C'est d'ailleurs jusqu'à cette échéance de 2027 que je vous propose de proroger le moratoire sur l'impératif

Parlement, en toute transparence et en responsabilité, de l'état d'avancement du programme immobilier pénitentiaire et de ses conséquences sur le taux de placement en cellule individuelle. Quatrièmement, je souhaite moderniser et agrandir l'immobilier juridictionnel. C'est indispensable si l'on veut accueillir les renforts humains qui sont attendus dans les années à venir. 502 millions d'euros d'autorisations d'engagement et 269 millions d'euros de crédits de paiement immobiliers sont prévus en 2023. Ces crédits permettront en outre de poursuivre les opérations majeures engagées lors du quinquennat précédent- je pense notamment aux palais de justice de Lille, de l'île de la Cité et de Bayonne -, de poursuivre -, de poursuivre l'étude des projets de Cayenne, Cussey, Meaux, Moulins, Nancy, Nantes, Perpignan, et de lancer de nouvelles opérations immobilières comme à Argentan, Chartres, Colmar, Saint-Brieuc ou encore Verdun. Cinquièmement, et enfin, permettez-moi de mettre en exergue certains efforts budgétaires. L'enveloppe de crédits consacrée aux dépenses de frais de justice sera portée à 660 millions d'euros, soit une hausse de 12 millions d'euros. Les crédits alloués aux investissements informatiques seront portés à 195 millions d'euros dans le cadre de la poursuite de la mise en oeuvre du plan de transformation numérique du ministère. Les crédits dédiés à l'aide juridictionnelle continueront de croître en 2023, pour atteindre 641 millions d'euros, soit une hausse de 26 millions d'euros en une année. Parallèlement, l'aide aux victimes sera portée à 43 millions d'euros, soit une hausse de 7

est à la croisée des chemins. Délaissé pendant près de trois décennies, son budget fait l'objet, depuis cinq ans, d'un renforcement massif de près de 4,7 milliards d'euros, traduction

en un claquement de doigts. La route est longue, bien sûr, mais j'espère que le Sénat, qui accorde à la justice une grande importance, à l'instar de ses commissions des lois et des finances, sera à nos côtés pour voter cette nouvelle hausse de 8

de l'article 5 de la loi

en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, intégrait un amendement rehaussant les crédits en faveur du dispositif téléphone grave danger, mais sans lever le gage. Dans mon rapport budgétaire, j'avais appelé le Gouvernement à lever ce gage, en rétablissant les crédits du programme « Justice judiciaire

Monsieur le garde des sceaux, les avocats nous confient que, dans près de la moitié des cas, leur rétribution au titre de l'aide juridictionnelle n'est pas suffisante pour couvrir les frais qu'ils engagent par dossier. Le rapport de la mission relative à l'avenir de la profession d'avocat, présidée par Dominique Perben, avait, à cet égard, recommandé de rehausser le montant de l'unité de valeur à 40 euros.

ce qui démontre votre grand attachement à la loi du chronomètre. Pourtant mes phrases restent raisonnables- je ne me compare pas à Marcel Proust, vous le savez bien. Vous eussiez donc pu me laisser finir ma phrase. Que disait la fin de la phrase ? Chacun s'interroge à ce sujet.

Mais il est possible, premièrement, de faire très attention aux courtes peines, qui ont souvent des effets négatifs, deuxièmement, de développer les alternatives à la détention, qui sont aussi des peines et qui sont efficaces, de travailler sur les aménagements de peine. De cela, vous n'avez nullement parlé, monsieur le garde des sceaux, dans votre propos introductif, mais j'espère que vous souscrirez à ces orientations, qui éviteront

Encore faut-il ensuite que les places soient occupées, mais cela relève moins de l'administration pénitentiaire que de la décision des magistrats. La diversification des postes a également tendance à s'accroître, ce qui ne peut être que positif pour l'insertion des détenus. La direction de l'administration pénitentiaire souhaite également redynamiser les partenariats

Le scrutin est clos.

qui ont perdu la pleine propriété et la possession de leur femme, continuent de développer leur vindicte à l'encontre de leur ex-épouse par l'intermédiaire des enfants.

de la même affaire. Elles s'attendent les unes les autres, chacune tenant l'autre en l'état, et les femmes sont coincées. Nous avons besoin de cette juridiction spécialisée.

par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

Je rappelle régulièrement, dans le cadre de mes travaux, qu'une politique pénitentiaire ne peut se résumer à une politique immobilière et à la construction de places supplémentaires en détention. Toutefois, et c'est là sans doute où nous divergeons, il me semble illusoire de croire pouvoir régler complètement la situation, à court terme, grâce un mécanisme de régulation carcérale.

vingt ans. Il permet d'accompagner et d'encadrer les personnes présentant un problème de santé mentale et ayant commis des infractions criminelles dans le processus judiciaire, tout en leur offrant les moyens d'améliorer leur situation. En France, les problèmes de santé mentale touchent huit fois plus de personnes dans la société carcérale que dans la société libre. Le présent amendement a ainsi pour objet de lancer une expérimentation dans le but de déployer le programme d'accompagnement justice-santé mentale en France.

prévention, même si cet enjeu mobilise au quotidien tous les services de l'État, notamment l'administration pénitentiaire.

la protection judiciaire de la jeunesse, un secteur en proie à une crise matérielle et des vocations depuis des années. Les crédits affectés au programme « Protection judiciaire de la jeunesse » se concentrent majoritairement dans la poursuite de création de nouveaux centres éducatifs fermés, très coûteux, sans remédier à la crise que subit le personnel de la PJJ.

Je ne suis toutefois pas d'accord sur le manque de moyens que vous mettez en avant, ni même sur la priorité qui serait donnée à la construction de centres éducatifs fermés. La hausse de 10,3 % des crédits alloués à la PJJ est en très grande partie tirée par l'augmentation des dépenses de personnel, qui s'explique par le relèvement du point d'indice, mais, surtout, par l'effet en année pleine des revalorisations décidées dans le cadre du Ségur.

En juillet dernier, la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté a dressé un constat accablant : le taux d'occupation global y était de 199 %, et même de 235 pour la maison d'arrêt des hommes ; 145 cellules étaient triplées avec un matelas au sol et de nombreux détenus avaient un espace personnel de moins de 3 mètres carrés. Dans la foulée, le 13 octobre dernier, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a enjoint au ministère de la justice de mettre en oeuvre neuf mesures, dont la rénovation des cellules. Cet amendement vise à ouvrir les crédits nécessaires à cette rénovation. Des mesures d'urgence doivent être prises, afin de garantir le respect des droits fondamentaux, d'autant que que le chantier de reconstruction de la prison, qui ne se terminera qu'en 2027, restera largement insuffisant, ces travaux permettant à peine d'absorber la surpopulation actuelle. Malheureusement, la prison de Gradignan n'est pas pas un cas isolé : en 2020, la justice française a alerté sur les conditions de vie indignes des détenus dans 35 établissements pénitentiaires. La France a également été condamnée à dix-huit reprises par la Cour européenne des droits de l'homme pour violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme En janvier 2020, cette même Cour européenne a condamné la France à prendre des mesures structurelles pour mettre un terme à la surpopulation carcérale.

négliger l'entretien et la rénovation de l'existant. Je vous communique donc les chiffres que j'ai obtenus : l'administration pénitentiaire disposera l'an prochain d'un budget inédit de 142 millions d'euros dédiés à la maintenance et à l'entretien des bâtiments. Ce montant est plus élevé que la moyenne de 110 millions d'euros

que les crédits nécessaires aux travaux d'amélioration de la prison de Gradignan sont inscrits dans l'enveloppe de rénovation des établissements, qui, je le rappelle,

Notre collègue insiste à juste titre sur l'équipement informatique et la numérisation des Spip. Je veux à cet égard rappeler que le plan de transformation numérique de la justice concerne l'ensemble des services et des métiers, y compris donc les Spip. Les crédits ne sont pas forcément labellisés sur ceux de l'administration pénitentiaire,

internet en prison. En 2020, la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté avait estimé dans un rapport que cet accès devait être considéré comme « prioritaire », considérant cette privation comme une « entrave » à de nombreux droits fondamentaux, dont la liberté d'expression, le droit à l'éducation et le droit d'une personne détenue à la préparation de son retour au sein de la société. La même année, la mission d'information du Sénat sur la lutte contre l'illectronisme et pour l'inclusion numérique qualifiait cette situation de « double peine » pour les personnes privées de liberté. Plusieurs pays ont d'ailleurs introduit des accès contrôlés

pour que l'on maintienne cette perspective de l'encellulement individuel, qui renforce bien entendu la dignité les conditions de détention et favorise

Si je suis donc d'accord pour dire que notre politique pénitentiaire ne doit pas se résumer à un programme immobilier, je suis hostile à la suppression de l'article, qui ne changera pas la situation.

en application de l'article L. 213-4 du code pénitentiaire. Si cette prorogation est nécessaire, elle n'en demeure pas moins un aveu des retards concédés par le Gouvernement en matière de politique pénitentiaire, cette dernière ne pouvant se résumer à la seule construction de places de détention supplémentaires. Par coordination avec le prolongement du moratoire, je propose au travers de cet amendement que le Gouvernement remette deux nouveaux rapports, en 2025 et 2027, ce qui permettra au Parlement de prendre connaissance, à intervalles réguliers, de l'exécution des programmes immobiliers pénitentiaires et de leur impact quant au respect de l'objectif de placement en cellule individuelle. l'avis du Gouvernement

je vous remercie souhaitées. Le Gouvernement a déjà engagé un travail sur l'évaluation de la charge de travail des magistrats. Il pourra peut-être nous indiquer s'il envisage de conduire la même démarche pour les autres métiers du ministère de la justice, qui sont eux aussi soumis à d'importantes tensions. La

Merci,